La séance est reprise. Nous poursuivons la discussion du projet de loi relatif à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires

le Parlement devra s'être prononcé sur le projet de loi de programmation sur l'énergie et le climat, qui fixera un cap et déterminera la planification censée en découler. Ainsi disposerons-nous d'une feuille de route qui devrait permettre de rebasculer dans les procédures normales de droit commun.

la période d'application des mesures du projet de loi relatives à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité des sites nucléaires existants. Actuellement, en effet, l'horizon des prévisions en matière d'énergie est fixé à

Cette disposition me paraît nécessaire pour assurer la bonne réussite du développement du nucléaire et, ainsi, améliorer la compétitivité de notre électricité et garantir la sécurité de notre approvisionnement.

qu'il s'agisse du périmètre, de la durée ou des types d'installation nucléaire concernés par les mesures de simplification et d'accélération des procédures de construction de réacteurs.

de la concertation avec l'ensemble des parties prenantes. Elle exige aussi une évaluation démocratique et pluraliste des besoins de notre société en matière d'énergie, dans un contexte de transition énergétique et de décarbonation de nos économies. Ce projet de loi, qui vise à accélérer les procédures pour amorcer la relance de la construction de nouveaux réacteurs nucléaires, ne saurait en aucun cas servir à anticiper sur les débats publics en cours et sur la future grande loi quinquennale que nous appelons tous de nos voeux.

Cet amendement vise à supprimer les électrolyseurs destinés à la production d'hydrogène du champ d'application du projet de loi,

soumis à la participation du public pour la construction de quatorze réacteurs pressurisés européens et de petits réacteurs modulaires. Cette démarche paraît prématurée dès lors que ce projet de loi porte sur la simplification des procédures et que les orientations, tant qualitatives que quantitatives, applicables au développement de nouveaux réacteurs nucléaires seront définies par le Parlement dans le prochain projet de loi de programmation sur l'énergie et le climat, que le Gouvernement prévoit de présenter dans les prochains mois. Le cadre approprié pour le suivi des projets qui en résulteront pourra alors être déterminé de manière cohérente.

La commission des affaires économiques a souhaité clarifier cette notion en se référant aux plans particuliers d'intervention. Les projets de réacteurs électronucléaires, aux termes de la rédaction issue des travaux de la commission, ne pourront être implantés que dans des zones n'excédant pas le périmètre du PPI. Toutes les installations

Par cet amendement, nous souhaitons un renforcement clair des garanties pour tous les travailleurs sous-traitants qui participent et participeront au déploiement de la filière électronucléaire. En 2009, nous alertions déjà sur les conditions de travail des travailleurs du nucléaire. Pour accroître la rentabilité des centrales et répondre à des injonctions financières contraires à la notion de service public et à la sûreté des installations, EDF et d'autres groupes publics du nucléaire ont recouru de manière massive à la sous-traitance pour la maintenance des installations, au point que, sur certains sites nucléaires, le personnel sous-traitant est devenu numériquement plus important que le personnel salarié d'EDF

Ce qui ressort de nombreux témoignages de salariés d'EDF ou encore d'Orano est sans appel : la sous-traitance nucléaire est massive et intervient dans tous les domaines- 80 % des activités de maintenance, la chimie de l'uranium, la gestion des déchets, le démantèlement.

ainsi que la collecte, le conditionnement et la gestion des déchets, mais aussi le montage d'échafaudages, le magasinage, la blanchisserie, et ce souvent de manière itinérante, de site en site, au rythme des « arrêts de tranche

Quel est l'avis de la commission ? Tout d'abord, les responsabilités sont déjà très bien définies par le code de l'environnement et le code de la santé publique. Une directive du 5 décembre 2013 fixe d'ailleurs aux États membres la nécessité d'établir les exigences légales et réglementaires. De plus, l'article L. 1333-7 du code de la santé publique oblige les responsables d'activités nucléaires à mettre en oeuvre les moyens et mesures permettant d'assurer la protection de la santé publique, de la salubrité et de la sécurité publiques, ainsi que de l'environnement.

amendement est donc déjà satisfait. Les relations de coactivité entre l'employeur de l'entreprise utilisatrice et les employeurs des entreprises extérieures sont, par ailleurs, réglementées par le code du travail, notamment par les articles R. 4511-1 et suivants. Pour toutes ces raisons, d'un point de vue technique et légistique,

de qualité des missions de service public. La grande entreprise qu'est EDF l'a d'ailleurs démontré depuis 1946. J'espère, madame la ministre, que le projet

et qui mettent en cause la sûreté des installations. Si notre filière nucléaire est aussi réputée, c'est qu'elle a été une filière d'excellence. Si nous voulons la relancer, il faut qu'elle le demeure,

Paoli-Gagin vise à prévoir que, dans les six mois suivant la promulgation de la loi, le ministre chargé de l'énergie expose devant le Parlement le calendrier opérationnel pour l'installation des futurs réacteurs nucléaires, conformément aux objectifs fixés par le Président de la République dans son discours de Belfort du 10 février 2022.

Si les ajouts du rapporteur tendent à améliorer sensiblement le dispositif, en prévoyant que la qualification de projet d'intérêt général (PIG) des nouveaux réacteurs n'interviendra qu'à l'issue du débat public organisé par la et en proposant une meilleure intégration des collectivités territoriales dans le processus de consultations préalables quant à la modification de leurs documents d'urbanisme, nous ne pouvons toutefois que demander la suppression de cet article. Nous nous opposons au principe même de la mise en place d'une procédure spécifique de mise en compatibilité des documents locaux d'urbanisme transférée en grande partie aux mains de l'État, au détriment des établissements publics de coopération Dans cette première phase du projet de construction, les collectivités territoriales concernées ainsi que leurs habitants se trouvent toujours bien trop marginalisés. Nous nous opposons à ce dessaisissement qui met à mal le principe de libre administration des collectivités territoriales. Enfin, les gains attendus de cette simplification abusive sont très exagérés. Elle ne fera gagner au projet que quelques mois, tout au plus. Ce ne sont pas les procédures d'instruction des demandes d'autorisations ou les procédures contentieuses engagées qui sont à l'origine de l'important retard des chantiers EPR en France et à travers le monde. Quel

Cet amendement vise à supprimer la précision introduite lors de l'examen du texte en commission, selon laquelle la qualification de projet d'intérêt général ne peut intervenir qu'à la condition de l'intervention préalable du bilan du débat public. Le droit en vigueur satisfait déjà cet Le droit en vigueur impose déjà d'attendre le bilan de la concertation avant de pouvoir prendre une décision de poursuite du projet. Cet amendement tend à clarifier la lisibilité du texte et ne porte pas atteinte à la participation du public. Il vise à sécuriser juridiquement la procédure. Par conséquent, le

communes ou des communautés d'agglomération.

: dans les faits, le département et la région seront informés très en amont, dès la fin du débat public, le porteur du projet de réacteur nucléaire devant publier un acte fixant les principes et les conditions de la poursuite de son projet. Le besoin de qualifier de projet d'intérêt général et de mettre en compatibilité des documents d'urbanisme sera identifié par cet acte. Encore une fois, je le rappelle, l'objet de ce projet de loi est de simplifier et d'accélérer les procédures

par l'État. Les services de l'État et les collectivités concernées peuvent dialoguer à n'importe quel moment de la procédure de mise en compatibilité sans qu'une étape obligatoire et contraignante soit formalisée. à de multiples reprises l'association de la collectivité concernée, que ce soit préalablement à la qualification du projet d'intérêt général, lors du débat public ou lors des concertations locales pour la mise en compatibilité du document d'urbanisme. La collectivité doit également nécessairement rendre son avis sur le projet de mise en compatibilité lors de l'examen conjoint et lors de la présentation du bilan de la participation du public. Le dialogue entre l'État et les collectivités est soutenu tout au long de la procédure. Nul besoin d'ajouter des étapes et de complexifier un processus ayant vocation à être

S'il y a urgence à créer des sites de production d'énergie nucléaire, y compris en agissant sur les sites existants, nous considérons qu'il ne faut pas ignorer tout le travail réalisé dans les communes et dans les intercommunalités pour accorder la priorité à certaines orientations, sanctuariser des espaces, définir une politique d'aménagement cohérente, avec des procédures d'élaboration et de modification des plans locaux d'urbanisme (PLU) qui peuvent être très longues et durer plusieurs années. Les échanges avec le public sont parfois source de critiques, mais ils permettent

durant lesquels les habitants des communes concernées pourront prendre connaissance dans le détail du projet de modification et s'exprimer.

Notre amendement vise à compléter le texte en précisant que la synthèse des observations et propositions du public, avec l'indication de celles dont il a été tenu compte, est rendue publique dans des conditions définies par arrêté.

que, lorsque la participation du public a lieu sous une forme dématérialisée, les populations devaient disposer d'un point d'accueil de proximité pour consulter sur support papier le dossier soumis à la consultation du public. Cet amendement vise à reprendre ce principe pour garantir un égal accès aux documents de la consultation, en prévoyant notamment la possibilité d'une consultation du dossier dans les préfectures et les sous-préfectures, la mairie du

du rôle des collectivités territoriales, d'autre part à retirer la mention du bilan des indications dont il a été tenu compte, puisque cette obligation serait impossible à remplir au vu du séquençage dans le temps de la procédure de mise en compatibilité.

Nous avons mesuré également le problème social posé par la sous-traitance. L'énergie nucléaire est une énergie d'élite. Pour autant, ses travailleurs doivent être traités avec davantage de dignité, ce qui n'est souvent pas le cas des sous-traitants- pour certains, qui viennent de l'autre bout de l'Europe et qui travaillent dans des conditions peu compatibles avec l'image de modernité qu'offre le nucléaire, et plus proches d'une version moderne de l'esclavage.

être très vigilant sur la responsabilité des donneurs d'ordre et leur faire appliquer la loi. C'est très exactement ce que nous souhaitons faire. Le Gouvernement

« l'ampleur, la complexité et la sensibilité d'un projet de création de centrale électronucléaire ». Nous estimons que cette dispense d'autorisation d'urbanisme n'est pas acceptable. Ce sont non pas les délais administratifs qui ralentissent la filière, mais bien l'instruction technique et le manque de compétences- parler des sous-traitances. La dérogation au droit commun n'est donc pas justifiée. Par ailleurs, le texte de la commission vise à exclure les emprises des futures centrales nucléaires du décompte des surfaces artificialisées au titre des objectifs du « zéro artificialisation nette cette nouvelle dérogation au respect des objectifs ZAN fixés par législateur ne nous paraît, pour le moins, pas justifiée. Cette disposition est symptomatique d'une tendance lourde de la droite sénatoriale, et très souvent du Gouvernement, qui est en totale contradiction avec les grandes promesses de verdissement celle du détricotage permanent du droit de l'environnement et du droit de l'urbanisme pour permettre des implantations toujours plus rapides de sites industriels, avec moins d'évaluation et de consultation du public. La préservation de la biodiversité au travers de la renaturation d'espaces artificialisés et la réduction de l'artificialisation des sols ne doivent pas être sacrifiées sur l'autel du développement de l'énergie nucléaire. Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à supprimer cet article. Quel

Cet amendement vise à rétablir la mention de l'autorité administrative, en lieu et place du ministre chargé de l'urbanisme, comme autorité compétente pour vérifier la conformité des réacteurs électronucléaires aux règles d'urbanisme applicables.

concernées, au regard des règles de droit, des enjeux et des caractéristiques locales propres à chaque territoire. Afin de garantir la meilleure prise en compte de ces caractéristiques, il est préférable de confier ce contrôle de conformité au représentant de l'État dans le département, qui dispose des compétences de toutes les administrations et d'une bonne connaissance du terrain. Quel est l'avis de la commission

sur le contenu du décret en Conseil d'État pris en application de l'article 3. D'une part, la rédaction actuelle de l'article 4 ainsi que les dispositions du code de l'environnement existantes permettent de satisfaire l'objectif de la commission sur ce point. D'autre part, il ne paraît pas utile de préciser le contenu de ce décret en Conseil d'État.

ministre. Il s'agit de clarifier le régime de fiscalité associé à la création des réacteurs électronucléaires. L'adoption de cet amendement permettra, d'une part, d'inclure un mécanisme dérogatoire concernant la taxe d'archéologie préventive similaire à celui qui est déjà prévu pour la taxe d'aménagement, d'autre part, d'améliorer la rédaction de de l'article 3, afin d'assurer la perception de ces taxes. Il s'agit également de clarifier le fait générateur de la taxe d'aménagement en prévoyant, comme c'était le cas dans la rédaction initiale de l'article, un fait générateur unique. la rédaction introduite en commission apporte un degré de complexité au calcul du montant de cette taxe, qui ne va pas dans le sens de la clarté du droit. Il est nécessaire de rétablir l'autorisation de création du réacteur électronucléaire, en application de l'article 596-7 du code de l'environnement, comme fait générateur de la taxe d'aménagement. Cette disposition permet ainsi de prendre en compte toutes les évolutions du projet pour le calcul du montant de cette taxe.

D'autre part, lors des auditions, nous avons entendu le message très clair des collectivités sur la taxe d'aménagement qui vise à compenser les coûts réels d'aménagement. Il ne faut donc pas réduire cette compensation, dont les retombées contribuent d'ailleurs de manière

une nouvelle installation nucléaire. Il s'agit d'adapter les délais d'autorisation pour plus de cohérence avec l'objectif d'accélération porté par le texte. Un délai d'instruction de douze mois semble raisonnable, tout en permettant un gain de temps non négligeable. Buis, pour présenter l'amendement n° 104 rectifié. Il est proposé de remplacer le décret en Conseil d'État actant l'autorisation environnementale par un décret simple sur la conclusion d'une instruction technique. Un décret en Conseil d'État ne paraît pas utile, en tout cas pas de nature à accélérer ou sécuriser davantage les projets de nouveaux réacteurs nucléaires.

car cette autorisation portera non pas sur les enjeux de sûreté nucléaire, mais plutôt sur les aspects préparatoires du chantier.

Il faut accélérer la production d'énergie nucléaire : nous voulons bien l'entendre, puisque, vous en conviendrez, mes chers collègues, nous soutenons cette idée depuis plusieurs années. Cependant, il est incompréhensible de considérer qu'avant d'être allé au bout des études, avant même d'avoir purgé tous les recours possibles, le porteur du projet pourrait lancer les travaux. 4 précise que le porteur assumera les risques, y compris financiers. Toutefois, quand le mal sera fait, on ne pourra pas le corriger en renvoyant nécessairement la faute sur le porteur de projet, à qui vous allez demander d'aller toujours plus vite, parfois au détriment du bon sens et à ses risques et périls.

M. Daniel Salmon. Il y a une incohérence manifeste à ce que des travaux concernant des « bâtiments annexes » puissent commencer à compter de la délivrance par décret de l'autorisation environnementale sur l'ensemble du projet et avant la clôture de l'enquête publique portant sur la création de la centrale. Si les modifications du rapporteur, qui introduisent des garanties relatives à l'évaluation environnementale et à la participation du public, vont dans le bon sens, cet amendement a pour objet la suppression de l'alinéa 2, qui permet le démarrage des travaux de construction des bâtiments annexes avant la délivrance de l'autorisation de création du réacteur. Les citoyens et les collectivités seraient mis encore une fois devant le fait accompli, puisque la centrale, dont l'enquête publique portera sur sa création, aura déjà commencé à être construite. Le gain de temps escompté, qui n'est d'ailleurs pas évalué, ne justifie pas une atteinte disproportionnée à la participation du public, sachant que les retards sont dus- on l'a dit et on le redit -aux difficultés industrielles et non administratives.

conditionnant le fonctionnement du réacteur électronucléaire. Omettre les équipements et installations, c'est se priver d'une partie opérationnelle de cet article, qui permet- je le rappelle -de démarrer certains travaux dès l'obtention d'une autorisation environnementale, donc, là encore, de gagner du temps. amendement tend à remplacer le ministre chargé de l'urbanisme par l'autorité administrative pour le contrôle des règles de fond d'urbanisme. Il se trouve que les autorisations ne relèvent pas

L'amendement n° 98 vise à tout supprimer. L'amendement n° 100 tend à ajouter de nouveaux équipements liés à l'exploitation des réacteurs et l'amendement n° 101 rectifié à retirer la référence au ministre chargé de l'urbanisme. Il ne me semble pas du tout opportun d'écarter ainsi le travail approfondi

la rédaction équilibrée de notre commission. Celle-ci vise simplement à garantir l'absence de difficultés sur le plan de la sûreté et de la sécurité et à rappeler les garanties légales applicables, dans un souci

une limite temporelle aux dispositions dérogatoires qui autorisent le Gouvernement à prendre, au début du projet, l'autorisation environnementale rendue nécessaire par les travaux de construction. Cela permet ainsi le retour au droit commun pendant l'exploitation du réacteur électronucléaire. Quel est l'avis de

de conserver la possibilité de modifier l'organisation à tout moment. Ensuite, le Gouvernement a clairement indiqué que les travaux afférents à l'autorisation environnementale, d'une part, et à l'autorisation de création, d'autre part, ne seraient pas effectués selon une logique séquentielle.

ainsi que l'intégration de nos installations électriques dans nos beaux paysages. Si j'ai bien compris notre collègue Gérard Longuet, la consultation publique n'a pas réellement d'importance dans nos choix énergétiques. Nous vous proposons ici de donner plutôt voix au chapitre aux maires dans la politique énergétique française. Il s'agit d'acter un principe simple : le droit de veto des communes visuellement touchées par l'implantation d'une centrale électronucléaire. La raison qui a prévalu au dépôt de cet amendement est paysagère : il s'agit de préserver la beauté des panoramas français. En effet, une centrale nucléaire est tout aussi dommageable, parfois plus pour certains, sur nos paysages qu'un champ d'éoliennes. Ceux qui ont déjà emprunté la vallée du Rhône peuvent témoigner que les centrales de Cruas ou du Tricastin ne valorisent pas cette belle vallée. Nous souhaitons donc, avec cet amendement, que les conseils municipaux des communes visuellement touchées par les nouvelles centrales puissent accepter ou non cette dégradation de leur qualité de vie.

lequel sont prévues un certain nombre de mesures relatives au système d'alerte en cas d'incident ou à la distribution de pastilles d'iode. C'est donc plus cohérent. Si les communes et leurs habitants sont touchés par ces mesures, il nous semble raisonnable que les conseils municipaux aient leur mot

: La parole est à Mme Monique de Marco. De nombreux territoires français sont menacés par un risque d'inondation ou de submersion marine. Dans l'estuaire de la Gironde, le trait de côte pourrait reculer de 479 mètres, selon les projections du Giec. Les conséquences sur nos installations nucléaires seraient majeures.

et sur un coefficient de marée de 120. L'inondation a endommagé le système de refroidissement et deux réacteurs ont été arrêtés en urgence. Je pense que personne ici ne souhaite revivre un tel événement. Ainsi, mes chers collègues, l'amendement que je vous propose d'adopter fait appel à votre bon sens : n'installons pas un réacteur nucléaire sur une zone vulnérable aux inondations et aux submersions marines. La catastrophe du Blayais a démontré notre incapacité à anticiper les conséquences des événements météorologiques majeurs. vrai que les modèles employés pour estimer ces risques comportent des failles et que les conséquences du dérèglement climatique demeurent imprévisibles. Au cours du siècle, la fréquence et l'intensité des catastrophes climatiques ne cesseront d'augmenter. Selon le Giec, la commune de Braud-et-Saint-Louis, où est implantée la centrale nucléaire du Blayais, devrait être régulièrement submergée. Par cet amendement, il s'agit tout simplement d'assurer la sûreté de notre parc nucléaire et la sécurité de nos concitoyens. monsieur le rapporteur,

ont choisi d'accorder de multiples dérogations en matière de rejets d'eau chaude dans les fleuves. Ces réponses administratives ne sont que des contournements qui permettent d'éviter soigneusement de se poser les bonnes questions sur la gestion de l'eau, sur les conflits d'usage et sur la préservation de la biodiversité en amont

Les épisodes extrêmes de sécheresse sont la preuve que le nucléaire est aussi vulnérable au changement climatique. Ainsi, mes chers collègues, à titre personnel, je voterai en faveur de cet amendement de bon sens. La parole est à M.

Cet amendement de simplification tend à réduire de dix-huit à douze mois la durée d'instruction d'une demande d'autorisation d'exploiter une nouvelle installation nucléaire. Il s'agit d'adapter les délais d'autorisation pour plus de cohérence avec l'objectif d'accélération

Vous proposez de réduire de dix-huit à douze mois le délai minimal entre le dépôt de la demande d'autorisation d'exploiter un réacteur, au titre du code de l'énergie, et sa mise en service. Or le droit applicable vise à imposer que l'exploitant dépose son dossier de demande d'autorisation d'exploiter au moins dix-huit mois avant la date maximale de mise en service du réacteur. En réalité, il s'agit d'une anticipation : plus vous fixez un délai délai qui l'oblige à être en conformité et à pouvoir obtenir son autorisation d'exploiter, plus vous engagez le projet sur un chemin critique.

entre les intérêts liés, d'une part, au développement économique et à l'aménagement du territoire, d'autre part, à la protection et à la mise en valeur de l'environnement. Le dispositif de cet article, contrairement aux dérogations très encadrées, actées dans le projet de loi relatif à l'accélération des énergies renouvelables, n'est pas une dérogation ponctuelle, assortie de conditions de procédure et de fond destinées à en encadrer l'usage, mais bien une dérogation de portée générale, même si son objet est limité aux nouvelles installations nucléaires implantées en continuité des sites existants. Le texte de la commission élargit la dérogation aux ouvrages de raccordement. Même si le dispositif est davantage encadré, la dérogation générale est toujours bien présente. Une dérogation, qui rompt brutalement l'équilibre des droits, porte également une atteinte disproportionnée à l'article 1 de la Charte de l'environnement, dès lors que, comme l'a récemment rappelé le Conseil constitutionnel, « la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ». Les dérogations aux règles environnementales ne sauraient s'appliquer que dans des circonstances exceptionnelles. Quel

de l'application de la loi Littoral les réacteurs nucléaires et leurs ouvrages de raccordement au réseau de transport d'électricité. Il s'agit d'installations compactes, en proximité des sites,

M. Daniel Salmon. La délivrance, à titre dérogatoire, de la concession d'utilisation du domaine public maritime nécessaire à la construction de nouveaux réacteurs nucléaires à proximité d'installations déjà situées en façade maritime à l'issue de l'enquête publique environnementale et sans déclaration d'utilité publique préalable ne nous semble pas justifiée. La commission a ajouté la référence à l'érosion côtière dans le cahier des charges des conditions d'utilisation du domaine public maritime. Mais une simple mention de la prise en compte de l'érosion côtière dans le cahier des charges de l'exploitant ne saurait pallier une information en amont du lancement des projets de construction sur la vulnérabilité des infrastructures au changement climatique. Cette vulnérabilité se manifestera de façon croissante du fait des bouleversements climatiques à venir, notamment avec la hausse du niveau de la mer pour les sites de Penly et Gravelines. Rien que dans l'estuaire de la Gironde, pour ce qui concerne Blayais, le trait de côte devrait reculer de 290 à 479 mètres, selon les projections du Giec. Les conséquences sur nos installations nucléaires seraient majeures. Par ailleurs, la disposition est beaucoup trop floue. Elle devrait préciser le type de démonstrations que l'opérateur est censé réaliser sur l'érosion côtière et porter sur le cycle de vie de l'installation, réacteur par réacteur. Les différents retours d'expérience d'accidents nucléaires devraient être obligatoirement pris en compte. Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

et Le Blayais sont situés en zone littorale. Le reste des réacteurs, qui en constituent la majorité, se situent dans des zones fluviales, aux abords des grands fleuves. C'est notamment le cas des plus puissants réacteurs, comme ceux de Civaux ou Chooz, d'importantes centrales, comme celle de Cattenom. Or les intempéries sont également susceptibles d'exposer ces sites à des crues, des inondations et d'autres risques liés au milieu aquatique. Afin de sécuriser l'implantation et l'exploitation des nouveaux réacteurs, il apparaît donc nécessaire d'étendre, au sein du cahier des charges des concessions, la prévention des risques de submersion, inondation et des risques liés à l'élévation des eaux aux réacteurs situés dans ces zones. Cet amendement vise donc à étendre, au sein du cahier des charges de la concession d'exploitation, la prévention des risques aux zones fluviales, sans préjudice des zones littorales déjà couvertes par le projet de loi.

Mme Angèle Préville. Les travaux de la commission ont permis de préciser le contenu du cahier des charges relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime qui seront accordées pour la construction de nouveaux réacteurs électronucléaires dans les zones littorales. Notre amendement tend à ajouter expressément les enjeux de préservation de la biodiversité et des écosystèmes à la liste des prescriptions s'imposant à l'exploitant. Les abords des sites nucléaires peuvent en effet présenter des enjeux de biodiversité importants. Cette connaissance de la biodiversité permet une gestion différenciée sur les sites de production, afin de concilier les enjeux écologiques et les enjeux industriels. Il est donc judicieux de l'inscrire dans la loi, afin d'entraîner une préoccupation effective, voire une vigilance La prise en compte de la biodiversité constitue déjà un enjeu majeur. Elle le sera aussi pour l'intégration et l'acceptation par les populations de nouvelles installations nucléaires, au sein des territoires qui les accueillent.

: La parole est à Mme Monique de Marco. Au cours du siècle, la fréquence et l'intensité des catastrophes climatiques ne cesseront d'augmenter. Les inondations, les submersions marines se multiplieront et le trait de côte reculera dans de nombreux territoires. Il est primordial de tenir compte de cette réalité au moment d'autoriser l'utilisation du domaine public maritime pour nos nouvelles installations nucléaires. Rappelons-nous l'inondation de la centrale nucléaire du Blayais, en Gironde, où les deux réacteurs ont été arrêtés d'urgence, à la suite d'un dysfonctionnement du système de refroidissement.

Si des précisions ont été apportées en commission pour mieux cibler les travaux entrant dans le champ de la procédure d'extrême urgence et pour appliquer les mêmes garanties que celles qui sont prévues pour les autres procédures d'expropriation, nous considérons cette dérogation pour acquérir de manière forcée certaines propriétés privées disproportionnée et injustifiée. Ce ne sont pas les procédures administratives ou les procédures contentieuses engagées contre les décisions prises qui sont à l'origine de l'important retard des chantiers EPR en France ; ce sont bien les capacités techniques de la filière du nucléaire. Une fois encore, on se trompe de cible, raison pour laquelle la suppression de cet article.

je souhaite maintenir le maximum de garanties pour

à l'exploitation ainsi que les ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d'électricité pour les mesures d'expropriation avec prise de position immédiate. L'accès au foncier est effectivement nécessaire pour garantir la faisabilité globale d'un projet et les réacteurs électronucléaires ne dérogent pas à cette règle. Je confirme que ces dispositions restent de dernier recours : ces mesures d'expropriation ne seront accordées que sous certaines conditions, qui feront d'ailleurs l'objet d'un avis conforme du Conseil d'État.

de plus précisé que, si des cas d'expropriation existent pour les postes, ils sont très rares pour les lignes, en raison des servitudes existantes. C'est pourquoi l'amendement n° 114, dont l'objet est d'étendre la procédure

Catherine Belrhiti. Disposer d'eau en abondance est l'une des conditions du bon fonctionnement des centrales nucléaires, principalement pour évacuer la part d'énergie thermique non transformée en énergie mécanique. Or ce besoin ne saurait se soustraire aux conditions d'une gestion vertueuse de nos ressources en eau, compte tenu de la raréfaction en raison du changement climatique, des épisodes de sécheresse et des tensions entre usages. Le rapport sur l'avenir de l'eau produit par la délégation à la prospective du Sénat a souligné l'existence de deux moyens de refroidissement des réacteurs, l'un étant plus vertueux que l'autre. Lorsque le réacteur est refroidi en circuit ouvert, le prélèvement en eau est très important. En aval du système de refroidissement, l'eau est restituée pratiquement en totalité au milieu, à une température supérieure à la température de l'eau lors de son prélèvement. Lorsque le réacteur est refroidi en circuit fermé, le prélèvement en eau est beaucoup plus modeste, de l'ordre de trente fois moins que dans le système précédent. Il en découle un usage nettement plus vertueux de nos ressources en eau. C'est donc cette méthode de refroidissement en circuit fermé qu'il faut favoriser

de M. le rapporteur. Je précise que l'enjeu dépend de l'emplacement du projet : en bord de mer, le sujet du circuit ouvert ne se pose pas

et que leur foncier mérite d'être mutualisé au titre de l'objectif ZAN, aussi est-il intuitif qu'une partie des recettes bénéficie à l'ensemble des collectivités territoriales et non aux seules collectivités d'implantation. Je rappelle, à cet égard,

Il est logique et souhaitable que les collectivités ou groupements d'implantation soient les premiers bénéficiaires de ces recettes fiscales. Par ailleurs, l'enveloppe nationalisée au titre de l'objectif zéro artificialisation nette, évoquée dans l'objet de l'amendement, n'existe pas encore.

nucléaire (IRSN). Or, depuis plusieurs années, l'ASN a vu sa charge de travail augmenter très fortement. Aux dossiers d'instruction classique se sont ajoutées de nouvelles demandes d'instruction autour des problématiques de prolongation des centrales nucléaires, démantèlement, saturation des piscines saturation des piscines de stockage ou phénomènes de corrosion. L'ASN et l'IRSN auront-ils suffisamment de moyens pour lancer de nouvelles études face à de nouveaux phénomènes imprévisibles, de nouvelles agressions naturelles, sans oublier les risques de cyberattaques ou les risques géopolitiques ? Pour toutes ces raisons, nous souhaitons qu'un audit recensant les besoins prévisionnels de l'ASN et de l'IRSN soit engagé, pour faire face à l'éventuelle relance du nucléaire dans un contexte marqué par l'incertitude. Cet audit s'appuiera sur les moyens techniques et humains du ministère de la transition énergétique, raison pour laquelle il n'est pas utile de gager l'amendement. Quel est l'avis de

sur la disponibilité des réacteurs au titre de la sécurité d'approvisionnement, au détriment de la sûreté. Les compétences de l'ASN et son pouvoir décisionnaire en sont encore amoindris, s'agissant des installations nucléaires dont la durée de vie technique dépasserait ainsi

Nous ne pouvons que nous y opposer. La décision de faire fonctionner la majorité des réacteurs au-delà de leur quatrième, voire de leur cinquième, visite décennale est lourde de conséquences pour la sûreté et la sécurité des installations

En cas de non-respect des prescriptions et des échéances, la commission des sanctions devra être saisie. L'amendement Les dispositions ajoutées par la commission des affaires économiques ont clarifié l'objet de l'enquête publique qui a lieu à l'occasion des réexamens des réacteurs nucléaires, après Toutefois, le texte de la commission renvoie au régime général des enquêtes publiques, alors que l'enquête publique dont il est ici question en diffère en plusieurs points. Ces adaptations ont été réalisées au niveau réglementaire par les articles R. articles R. 593-62-2 à R. 593-62-8 du code de l'environnement. La référence à l'article L. 593-9, concernant l'enquête publique sur la demande d'autorisation de création d'installation,

Pour autant, dans un esprit de compromis, je suis disposée à le retirer au profit de la proposition du rapporteur contenue dans l'amendement n° 130, lequel tend à apporter une ouverture sur les adaptations réglementaires pour prendre en compte les spécificités de cette enquête publique de prolongation, qui ne saurait être assimilée à l'enquête publique initiale de création d'installation.

complémentaires conditionnant la poursuite de l'exploitation, ou de proposer au Gouvernement une mesure de mise à l'arrêt définitif d'installations inexploitées pendant plus de deux ans. Le principe de cette délégation technique et administrative est légitime, mais le Parlement pourrait mieux préserver son rôle de contrôle en qualifiant davantage cette délégation à une autorité administrative indépendante. L'adoption de prescriptions additionnelles de sûreté nucléaire pour autoriser la poursuite d'exploitation des réacteurs après quarante ans ne peut se concevoir à travers les seuls filtres de la technique réglementaire, des connaissances scientifiques et des technologies effectivement disponibles. Il faut également prendre en compte les attentes et les contraintes de la société au sens large, qui a besoin de sûreté, mais aussi d'accès à l'énergie électrique.

de disposer d'un fondement solide pour ses propositions, et aux autorités nationales compétentes- Gouvernement, Parlement, Cour des comptes ... -de mieux apprécier le bien-fondé desdites propositions.

l'exploitant a déjà l'obligation de transmettre annuellement un bilan des actions mises en oeuvre. Cet amendement tend aussi à revenir sur les dispositions concernant les modifications issues du réexamen. La commission des affaires économiques a introduit dans le texte une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire fixant la liste des modifications soumises à déclaration

Sans entrer dans le détail, une fois encore, dans un esprit de compromis, nous sommes prêts à retirer cet amendement du Gouvernement au profit de l'amendement n° 131 de M. le rapporteur. je propose que nous poursuivions, dans la suite de la navette parlementaire, les travaux de simplification de ce processus de réexamen pour en éliminer les étapes formelles superflues, afin que les acteurs du secteur se concentrent sur le fond : la sûreté et la performance de leur installation.

M. Daniel Salmon. Cet amendement vise à renforcer le dispositif prévu à l'article 9 ajouté en commission. Le changement climatique et le vieillissement des centrales imposent une vigilance accrue quant à la sûreté du nucléaire.

des réacteurs nucléaires existants, notamment de ceux qui sont engagés dans le programme de grand carénage. En cohérence avec nos positions précédentes concernant le périmètre du texte, il n'y a pas lieu, à nos yeux, de revoir le régime des autorisations d'urbanisme relatives aux travaux nécessaires au fonctionnement et à la mise à niveau des installations nucléaires existantes.

et à la protection de l'environnement. Une telle situation conduirait donc à considérer que les conditions posées à la délivrance de l'autorisation initiale ne sont plus satisfaites. Derrière le paravent de l'accélération, on favorise ainsi une pression sur la disponibilité des réacteurs au titre de la sécurité de l'approvisionnement, au détriment

Salmon. Cet amendement reprend l'article 10 de notre proposition de loi portant diverses mesures visant à renforcer la sûreté nucléaire, la transparence financière et le contrôle parlementaire. Afin d'assurer autant que possible une gestion responsable et raisonnée des déchets nucléaires, cet amendement vise à faire évoluer la doctrine entourant les matières radioactives que l'industrie nucléaire stocke en vue d'une hypothétique valorisation et qui représentent de nombreux déchets en devenir. Il importe que les données et les informations sur le retraitement des combustibles usés et sur les aspects techniques, économiques, financiers et environnementaux de la gestion des matières et déchets radioactifs et de leur valorisation soient renforcées. Rappelons que les opérations d'aval du cycle représentent environ 10 % du coût de production de l'électricité nucléaire.

De même, la question des critères de valorisation des matériaux nucléaires, dont la requalification aurait pour conséquence d'augmenter significativement les coûts de gestion des déchets, doit être clarifiée par la loi. Il nous paraît primordial d'éclairer le débat public, et en premier lieu le législateur, afin d'orienter les choix scientifiques qui engageront collectivement le pays. Tel est l'objet de cet amendement, qui reprend l'article 9 de notre proposition de loi. Nous souhaitons donc disposer d'un rapport d'évaluation des coûts de chacune des pistes

Ces installations nucléaires sont vulnérables et présentent des risques majeurs pour la sécurité de nos concitoyens. Or les modèles employés pour estimer ces risques comportent des failles et les conséquences du dérèglement climatique demeurent imprévisibles. La catastrophe du Blayais, en 1999, nous rappelle que la menace est constante. Aussi cet amendement vise-t-il à renforcer la sûreté de notre parc nucléaire en fermant les installations les plus vulnérables aux inondations et aux submersions marines. les dispositions contenues à l'article L. 593-23 du code de l'environnement, lequel prévoit la fermeture des installations présentant des risques graves pour la sécurité et la santé de nos concitoyens.

sens, le minimum de transparence que l'on peut exiger d'une filière qui, pendant quarante ans, a fonctionné comme un État dans l'État et a conduit EDF à la faillite. Nous avons suffisamment souffert de cette collusion entre EDF, l'administration centrale et le pouvoir exécutif, pour le résultat désastreux dont on fait le constat sur toutes ces travées. Il est temps de s'appuyer sur l'intelligence collective du Parlement pour engager les choix stratégiques du pays et assurer la sécurité de nos concitoyens. Nous ne Nous ne comprendrions pas que des parlementaires si désireux de participer aux choix stratégiques de la Nation en matière énergétique ne votent pas cet amendement. Quel

La loi du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs a créé une Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs (Cnef) ayant pour mission de vérifier l'adéquation des provisions aux charges. Cette commission peut demander aux exploitants communication de tout document nécessaire à l'accomplissement de ses missions et entendre l'autorité administrative qui instruit les dossiers. La Cnef s'est réunie pour la première fois le 17 juin 2011, soit près de cinq ans après la publication de la loi. Quelle célérité ! Elle a remis son unique rapport en juillet 2012. Depuis, ses activités ont cessé. À la suite des travaux menés en 2016 et 2017 par la mission d'information de l'Assemblée nationale sur la faisabilité technique et financière du démantèlement des centrales nucléaires, la commission d'enquête sur la sûreté et la sécurité des installations nucléaires créée le 1 février 2018, dont la rapporteure était la députée Barbara Pompili, a constaté que le provisionnement pour charge de démantèlement réalisé par EDF se révèle largement « illiquide largement « illiquide ». Elle a considéré qu'il ne peut revenir à l'exploitant, juge et partie, de fixer le montant des sommes à provisionner. Il conviendrait de s'inspirer du modèle de la commission des provisions nucléaires instituée en Belgique en 2003, qui a fait ses preuves.

que ce dernier dispose de toutes les informations nécessaires, notamment financières, pour orienter les choix scientifiques qui engagent collectivement tout un pays. Sur le sujet essentiel du nucléaire, les perspectives temporelles et l'étendue des sommes en jeu doivent mobiliser le législateur financier d'impulser l'obligation de transparence de la puissance publique. C'est ce qui a été fait, par exemple, à l'article 135 de la loi de finances du 29 décembre 2015 pour 2016, qui a imposé un rapport sur le financement des commissions locales d'information nucléaire, ou à l'article 90 de la loi de finances du 29 décembre 2014 pour 2015, qui a imposé un rapport sur le financement

Le président-directeur général d'EDF de 2014 à 2022, M. Jean-Bernard Lévy, a laissé entendre que l'entreprise travaillait sur un programme de fermeture échelonné sur une trentaine d'années, entre 2029 pour les premiers réacteurs qui seront arrêtés après cinquante ans d'exploitation, et 2060 pour les derniers réacteurs menés à soixante années d'exploitation. effort de transparence soit consenti afin de publier un échéancier prévisionnel approximatif des réacteurs à fermer, et donc à démanteler à ces deux échéances, dans le but de donner de la visibilité aux industriels concernés, aux salariés travaillant sur les sites ainsi qu'aux territoires qui doivent se préparer à l'après-nucléaire. Enfin, il apparaît que la filière nucléaire pourrait manquer de ressources humaines au cours des années à venir. Le secteur aura encore, et pour longtemps, besoin d'ingénieurs, de techniciens et d'ouvriers pour mener à bien l'énorme chantier du démantèlement. Une main-d'oeuvre importante sera également nécessaire pour prolonger l'activité des réacteurs qui ne seront pas immédiatement arrêtés. Un véritable travail prospectif doit donc être engagé pour évaluer les besoins en formation pour les années à venir, aussi bien pour développer la filière du démantèlement que pour la prolongation de certains réacteurs. Cet

de la centrale de Zaporijia, nous rappelle qu'un accident nucléaire par agression externe n'est pas à exclure. Le code de la sécurité intérieure prévoit que les plans d'organisation de la réponse de sécurité civile (Orsec) définissent un plan particulier d'intervention lorsqu'il existe des risques de nature particulière ou liés à l'existence et au fonctionnement d'installations ou d'ouvrages déterminés. En ce qui concerne les centrales nucléaires, les PPI permettent d'organiser la prévention, l'alerte et le secours aux populations en cas d'accident nucléaire. En France, le périmètre des PPI, fixé par l'État à vingt kilomètres autour de l'installation, conditionne la distribution de pastilles d'iode, qui réduisent le risque de cancer et de troubles de la thyroïde après une exposition radioactive. Chez nos voisins directs, ce périmètre est bien plus étendu- il est de quarante kilomètres

limites administratives. Plus encore, si cette disposition a été présentée dans le cadre d'une proposition de loi, je rappelle que, depuis lors, les PPI ont été étendus de dix à vingt kilomètres,